La séance est reprise. Mes chers collègues, mercredi 31 janvier, en raison de la tenue de la conférence des présidents à dix-neuf heures et en accord avec le groupe Les Républicains, les commissions concernées et le Gouvernement, l'examen de la de la suite éventuelle de la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux, puis l'examen de la proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public commenceraient à vingt Par ailleurs, il sera procédé au dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes jeudi 8 février, à dix heures trente. Y a-t-il des observations ? ? ... Il en est ainsi décidé. Enfin, le groupe Union Centriste a demandé de limiter à quarante-cinq minutes la durée de la discussion générale sur la proposition de loi créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap examinée au sein de son espace réservé du mercredi 31 janvier 2018. Acte est donné de cette demande.

Il faut faire des réformes. Il faut envisager, par exemple, une réorganisation de l'entreprise. Il faut envisager de modifier le système des régimes spéciaux. Il faut envisager une réforme du statut. Il faut envisager une réforme du rythme même des rotations. » Vous allez conclure que la droite veut déclarer la guerre à la SNCF. Manque de chance, ce sont les déclarations du Président de la République

bien compris que vous vous interrogiez sur l'ouverture à la concurrence, et c'est vrai que c'est un problème compliqué. Mais nous allons aider l'entreprise, et vous allez voir ce que vous allez voir : dans cinq ou six ans, l'entreprise SNCF sera prête à l'ouverture à la concurrence

à la direction de la SNCF ? Personne ne remet en cause les traditions de cette entreprise publique. Tous les Français sont très attachés à leur entreprise ferroviaire. Mais il ne faut pas la laisser mourir sous la dette,

je vous ai écouté attentivement. Je partage certaines de vos interrogations et de vos préoccupations, mais pas nécessairement tous vos propos. Personne dans cet hémicycle ne nie les dysfonctionnements qui ont eu lieu ces derniers mois. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur les événements survenus à la gare Montparnasse l'été dernier ou à Bercy à Noël,

qui m'ont présenté leur nouveau plan de management des travaux qui vont intervenir sur le réseau, travaux qui sont une des causes de dysfonctionnement ; ils vont également engager un audit des grandes gares du pays.

l'État a sa part de responsabilité, avec un sous-entretien et un sous-investissement dans les réseaux existants, en lien avec une politique du tout-TGV

Mais investir plus de 5 milliards d'euros dans le réseau- ce qui est une bonne nouvelle, puisque cela signifie investir pour des infrastructures rénovées et plus efficaces, investir dans l'avenir et dans l'outil de production de la SNCF -engendrera, vous l'imaginez, des désagréments temporaires, car il faudra bien réaliser les travaux. Personne ne peut affirmer aujourd'hui

C'est pourquoi j'ai également demandé aux opérateurs d'être particulièrement vigilants quant à l'information des voyageurs, lorsque la situation est perturbée. Je partage ici vos préoccupations : il n'est pas acceptable que les Français ne puissent pas bénéficier d'une information claire, simple et efficace sur les possibilités de déplacements qui s'offrent à eux. Cependant, on ne peut pas évoquer uniquement les trains qui n'arrivent pas à l'heure ; je souhaite ici, devant vous, saluer le formidable investissement des agents de la SNCF et leur volonté quotidienne d'offrir aux Français les meilleures conditions de transport. Alors que la SNCF célèbre ses quatre-vingts ans d'existence en 2018, le trafic a atteint en 2017 des records, qui sont la preuve de l'attachement des Français au transport ferroviaire. En 2017, la fréquentation a progressé de 10 % dans les TGV, de 8 % dans les Intercités- je rappelle que l'État

en région parisienne. Cette croissance du trafic est également la preuve que la santé économique du pays s'améliore, car, quand la croissance est là, elle engendre plus de trafic, ce qui est un bon signe.

je souhaite que le TGV soit populaire et accessible à tous. Nous avons fait un choix collectif depuis toujours d'avoir des TGV qui vont partout, au-delà du réseau à grande vitesse.

mon devoir en tant que ministre chargée des transports n'est pas uniquement de faire en sorte que tout aille mieux en 2018. C'est aussi de prévoir l'avenir pour projeter la France et son modèle ferroviaire dans le XXI siècle ; je veux rappeler ma détermination sur ce point. L'État se dotera dès cette année d'une stratégie claire pour le ferroviaire. C'est le sens des missions confiées à Jean-Cyril Spinetta pour une réflexion d'ensemble sur le modèle ferroviaire.

Au vu de ces deux rapports qui seront rendus à la fin du mois, le Gouvernement proposera une stratégie ambitieuse. Au printemps, nous aurons à débattre du modèle ferroviaire et d'une programmation soutenable. Car nous devons collectivement redéfinir ce que notre pays attend de ses trains, remettre le modèle économique en état de marche- 3 milliards d'euros de dette par an, ce n'est pas soutenable -et réussir l'ouverture à la concurrence prévue par les textes européens et demandée par les régions, c'est-à-dire plus de voyageurs dans les trains, une plus grande satisfaction des clients, un meilleur rapport qualité-prix et des cheminots rassurés sur leur avenir. Ma méthode est simple. Elle repose sur la concertation avec l'ensemble des acteurs. J'en veux pour preuve le succès des Assises nationales de la mobilité. Préparer les mobilités des prochaines décennies, c'est-à-dire la mobilité pour tous et dans tous les territoires, est un véritable projet d'aménagement du territoire. Nous travaillerons donc avec tous les élus, ainsi qu'avec les régions et les agglomérations. Selon les choix qui seront faits, des investissements seront bien sûr réalisés. Mais il faut que nous tirions le meilleur parti de chaque solution. Le TER doit aussi être un transport de masse, avec davantage de voyageurs dans les trains. Je pense que le ferroviaire doit jouer un rôle plus important dans nos agglomérations. Je tiens à le redire devant vous, une politique de mobilité ne se résume pas à une politique d'infrastructure. C'est tout l'esprit des Assises de la mobilité. Je pense à notre formidable capacité à innover, et je souhaite que nous puissions inventer de nouvelles réponses aux besoins de déplacements, qu'il s'agisse de véhicules autonomes, de covoiturage ou encore de l'ouverture des données. Concernant la SNCF et son avenir, je le dis très sereinement, j'ai confiance dans le modèle ferroviaire français, dans sa capacité à évoluer et à se moderniser. J'ai confiance dans le regard que portent les Français sur leur opérateur historique et dans les agents qui y travaillent au quotidien. Nous aurons l'occasion au printemps de discuter ensemble dans un esprit constructif de définir conjointement les grandes orientations du modèle ferroviaire de demain, pour les territoires que vous représentez et pour la Nation tout entière.

Le système actuel de redevances date de 2008 et le niveau des péages aujourd'hui constaté, vous l'avez souligné, est le fruit d'évolutions successives qui ont obéi à des logiques budgétaires et peu prévisibles. En conséquence, les tarifs sont peu justifiés et manquent de lisibilité pour les opérateurs. Cette refonte tarifaire est obligatoire pour mettre en conformité les barèmes des péages avec les règles européennes qui imposent une tarification « au coût direct », c'est-à-dire au prix permettant de couvrir le coût lié à la circulation d'un train, ce qui n'est pas le cas de la redevance de circulation facturée aujourd'hui aux TER et aux trains de fret. Pour couvrir, au-delà du « coût direct », tout ou partie des coûts fixes du réseau, les majorations tarifaires doivent être justifiées. Le déséquilibre persistant de la situation financière de SNCF Réseau est bien évidemment une réalité qu'il importe d'intégrer. Pour autant, ce déséquilibre ne saurait détourner le gestionnaire de l'infrastructure d'un objectif indispensable de la réforme ferroviaire : rétablir de bons signaux économiques incitant à optimiser l'utilisation du réseau et à rationaliser les choix d'investissement. Ce sont plus de 5 milliards d'euros qui seront engagés cette année dans le cadre des 1 700 chantiers programmés sur le réseau pour l'année 2018. SNCF Réseau est ainsi dans son rôle, mais doit aussi composer avec une dette abyssale de plus de 45 milliards d'euros. Voilà autant de freins incompressibles pour imaginer que la situation évolue favorablement ; il est donc essentiel que l'État puisse être à la manoeuvre pour imaginer des solutions permettant de sortir de cette spirale infernale. Madame la ministre, pouvez-vous nous en dire plus sur les pistes aujourd'hui imaginées pour sortir de cette impasse financière ? La

en réduisant les déficits annuels de SNCF Réseau et en revenant à l'équilibre, est un sujet majeur de préoccupation pour le Gouvernement. Au demeurant, l'Europe nous interroge également. se trouve au coeur du contrat entre l'État et SNCF Réseau, qui prévoit une stabilisation de la dette à l'horizon de 2026 à un niveau de 63 milliards d'euros, soit largement au-dessus des 50 milliards d'euros que nous atteindrons cette année. Les efforts prévus dans le cadre du contrat sont également complétés par le dispositif dit de la « règle d'or », qui interdit à SNCF Réseau

infrastructures, participer financièrement aux investissements de développement. Par ailleurs, si la trajectoire du contrat constitue aujourd'hui une référence, les réflexions sur l'assainissement financier de ce secteur doivent se poursuivre. En particulier, les hypothèses très dynamiques de péage retenues posent question au regard de leur soutenabilité par les entreprises ferroviaires. La mission confiée à Jean-Cyril Spinetta vise à porter un regard d'ensemble sur le modèle économique du ferroviaire et à interroger les hypothèses sous-jacentes à ce contrat. Dans ce cadre, la question du traitement de la dette historique de SNCF Réseau sera nécessairement posée.

La privatisation du rail imposée par Bruxelles et présentée par beaucoup comme l'ultime solution n'est pas souhaitable si l'on veut conserver un véritable service public pour tous. Le ferroviaire est un élément tellement indispensable à la lutte contre le réchauffement climatique qu'il est aberrant que la puissance publique se dessaisisse de ses prérogatives stratégiques sur le rail. On oublie de rappeler que les pays qui sont souvent cités en exemple de la libéralisation- la Suède, l'Allemagne -subventionnent par ailleurs très largement leur réseau ferré et ont mis en place une véritable politique de développement du rail- voyageur ou fret -sur leur territoire. J'ai déjà eu l'occasion de saluer les choix du Gouvernement de suspendre certains grands projets de lignes à grande vitesse pour réorienter une partie des financements vers le réseau secondaire, comme vous l'avez rappelé, ce réseau régional de proximité si essentiel qui fait au quotidien la vitalité de nos territoires. C'est le cas, notamment, de l'étoile ferroviaire de Veynes, seule liaison ferrée entre le nord et le sud du massif alpin. Mais, comme de nombreuses autres à travers le pays, cette ligne, faute de financements suffisants, se dégrade lentement et perd des usagers à mesure qu'elle perd en qualité, s'enfermant dans un cercle vicieux. Les régions, qui ont fourni un effort considérable pour préserver le ferroviaire régional, subissent aujourd'hui des baisses de dotations, ce dont pâtit grandement le réseau. SNCF Réseau, propriétaire des lignes et bénéficiaire des péages ferroviaires, ne finance plus les travaux de rénovation qu'à hauteur de 15 % de leur montant. L'argent collecté par les péages n'est plus totalement réinjecté sur l'entretien des lignes. Les régions se retrouvent dans la situation d'un locataire dans l'obligation de prendre à sa charge les travaux de rénovation de son appartement en lieu et place du propriétaire défaillant. Une nouvelle organisation est à envisager pour ces lignes locales. Si la « régionalisation » est une piste, notamment en ce qui concerne l'exploitation, elle ne doit pas se traduire par un désengagement complet de l'État.

Mme la ministre. Monsieur le sénateur, la ligne que vous mentionnez est en effet une des illustrations des défauts d'entretien et d'investissement qu'a connus notre réseau, je le redis, au cours des dernières décennies.

sur les meilleures modalités pour faire face à cette situation et pour répondre aux besoins de nos concitoyens, avec un objectif clair : maintenir une accessibilité dans ces territoires, quel qu'en soit le mode. Depuis 2009, l'ARAFER doit formuler des avis sur les conditions d'accès aux infrastructures ferroviaires : des avis juridiquement contraignants sur les tarifs et des avis consultatifs sur les conditions techniques et contractuelles. le décret du 7 septembre 2017, le Gouvernement est venu au secours de SNCF Réseau, qui faisait face à un avis défavorable de l'ARAFER en matière de tarifs. Ce décret supprime le caractère « juridiquement contraignant » de l'avis de l'ARAFER sur SNCF Réseau et permet à celle-ci d'augmenter ses prix au détriment des opérateurs et, par conséquent, des usagers et des régions. Le Gouvernement a ainsi assoupli le contrôle de l'ARAFER, et ce contre l'avis, entre autres instances, du CNEN, représentant les collectivités territoriales, en particulier les régions. Le 8 janvier dernier, vous avez souligné, madame la ministre, la nécessité de conduire un audit au sein de SNCF Réseau ... Ce qui se comprend bien, parce qu'avoir supprimé le caractère contraignant des avis de l'ARAFER sur SNCF Réseau pose clairement un problème pour s'assurer que l'entreprise respecte bien ses engagements contractuels à l'égard de l'État. Comment en sortir ? On ne voit pas bien en quoi un énième audit réglera la question. Madame la ministre, envisagez-vous de revenir sur le décret du 7 septembre 2017 ou, à défaut, de confier à l'ARAFER les moyens de s'assurer que SNCF Réseau respectera bien ses engagements contractuels ?

a effectivement prononcé un avis défavorable sur le projet de tarification pour 2018 soumis par SNCF Réseau en soulevant des questions de fond sur la structuration des péages, sur la nature des coûts à répercuter et sur la prise en compte du marché, comme le permet la réglementation européenne. Il n'est pas apparu possible, en l'espace des quelques semaines dont disposait le Gouvernement, de revoir en profondeur les principes de tarification applicables pour l'année 2018. C'est dans ce contexte qu'un décret a permis d'assurer une simple indexation de la tarification qui existait en 2017. Pour 2019, le projet de tarification a été adopté par le conseil d'administration de SNCF Réseau le 30 novembre dernier. Il est actuellement soumis à l'avis conforme de l'ARAFER, qui rendra ses conclusions début février. L'ARAFER, comme je l'ai souligné, a souhaité un meilleur reflet des coûts. C'est ce qui est intégré dans le projet de tarification pour 2019, lequel, sans entrer dans des détails trop techniques,

compte de la possibilité offerte de tarifer au-delà du coût marginal si le marché s'y prête. Cette nouvelle tarification suppose une adaptation du cadre réglementaire. C'est pourquoi un décret revoyant la structure de la tarification, en lien avec les demandes de l'ARAFER, a été préparé par le Gouvernement. Il sera très prochainement soumis à l'avis de l'ARAFER pour disposer d'un cadre répondant aux enjeux économiques de SNCF Réseau et respectant à la fois les principes fixés par la loi et

L'ouverture prochaine à la concurrence, conformément aux règles européennes, n'est pas sans susciter de vives inquiétudes chez les salariés du groupe SNCF. Certains pointent le risque lié à un manque d'anticipation et dénoncent l'absence de cadrage précis des conditions de cette ouverture. Deux thématiques sont principalement mises en avant. La première est relative aux périmètres concernés par cette ouverture. Ils doivent en effet être strictement définis et leurs impacts évalués sur le plan économique, social et fonctionnel, et ce préalablement au lancement de chaque appel d'offres. Il semble également, afin de ne pas déstabiliser le système, qu'une progressivité dans l'ouverture de ces appels d'offres serait nécessaire. La seconde thématique concerne bien évidemment les personnels, qui souhaitent, en cas de transfert, une garantie sociale assurant aux agents de la SNCF le maintien du statut et des droits qui y sont associés. la mise en place d'une garantie de l'emploi pendant la durée du marché. De même, la création d'un droit au transfert avec option du salarié, permettant ainsi aux agents de choisir leur avenir, est souvent évoquée. Ce dernier point me semble d'ailleurs fondamental, témoignant ainsi de l'attachement de bon nombre de cheminots au groupe public ferroviaire en dépit des mobilités géographiques qu'il imposera pour ceux qui choisiraient de rester au sein du groupe.

Mme la ministre. Monsieur le sénateur, l'ouverture à la concurrence, si elle n'est pas une surprise, est néanmoins une transformation profonde que nous devons préparer et discuter avec l'ensemble des parties prenantes, qu'il s'agisse des autorités organisatrices régionales ou, bien sûr, des cheminots. C'est le sens de la mission qui a été confiée à Jean-Cyril Spinetta.

une forte implication de la Nation dans la mise à niveau de notre modèle économique, avec une ouverture à la concurrence

Des améliorations sont nécessaires. La SNCF en est consciente. Pour ce faire, elle a déjà pris des mesures, notamment avec le programme ROBIN. Les critiques formulées en France, il faut le savoir, ont des conséquences sur l'exploitation du groupe à l'international. Or, la SNCF, ce ne sont pas que des retards. Ce sont 14 220 trains sur le réseau par jour, avec un taux moyen de ponctualité de 88 % pour le Transilien, de 89 % pour les TGV et de 91 % pour les TER.

J'ai siégé pendant plusieurs années au conseil d'administration de RFF, qui a poursuivi les dossiers déjà engagés par la SNCF. J'ai pu me rendre compte du rôle de l'État dans la définition des stratégies du groupe et des considérations parfois étrangères à l'intérêt général. Si, aujourd'hui, il y a des pannes et des retards, c'est en partie la faute de l'État et des politiques de tous horizons, qui ont préféré investir dans les LGV plutôt que dans la rénovation du réseau. un exemple parmi d'autres, à savoir le projet de LGV Poitiers-Limoges. Initié par Jacques Chirac, le projet a été relancé par François Hollande en 2016 après que le Conseil d'État eut pourtant jugé illégale la déclaration d'utilité publique. En plus de dix ans, le coût des études de ce projet à l'arrêt s'élève à près de 200 millions d'euros pour une voie

pour remettre à niveau notre réseau. C'est bien le sens du diagnostic qui a été lancé par SNCF Réseau pour anticiper les points de fragilité dans les grandes gares, qu'elles soient parisiennes ou en région,

Madame la ministre, j'ai lu avec attention le compte rendu de votre entretien avec Guillaume Pepy, PDG de SNCF Mobilités, et Patrick Jeantet, PDG de SNCF Réseau, à la suite des dysfonctionnements qu'ont connus les grandes gares parisiennes ces derniers temps. Vous avez annoncé que 5,2 milliards d'euros seront consacrés dès 2018 à l'entretien et à la régénération du réseau, lequel a souffert d'un sous-investissement dramatique depuis plusieurs décennies en raison des sommes très importantes mobilisées par la construction des lignes à grande vitesse, mais nous aimerions connaître le fléchage de ces financements. Vous le savez, l'état de nombreuses lignes d'irrigation du territoire est lui aussi globalement mauvais. Or ces lignes sont absolument indispensables au désenclavement de nos départements ruraux. Je prendrai l'exemple de mon département, le Cantal, l'un des plus enclavés de France. C'est vrai ! La ligne Aurillac-Clermont risque de connaître une réduction de vitesse à 60 kilomètres par heure sur certaines portions du trajet si des travaux ne sont pas réalisés rapidement. La ligne Aurillac-Brive, qui ouvre le Cantal vers l'ouest, pourrait, quant à elle, connaître une suspension d'exploitation en 2021 si les 20 millions d'euros nécessaires ne sont pas débloqués. Nos temps de trajet pour rejoindre Paris se sont rallongés- cinq heures trente en -et nous ne disposons d'aucun train direct, ce qui représente une vraie régression. La gare de Saint-Flour est en sursis. Vous le voyez, la situation du Cantal est absolument dramatique. Ma question est donc simple : la régénération de ces petites lignes, essentielles à la vie de notre ruralité, est-elle bien budgétée dans les 5,2 milliards d'euros des travaux est urgente, indispensable pour que nous puissions sortir de chez nous et y revenir, et surtout pour donner corps à l'égalité des citoyens devant le service public et favoriser le développement de nos territoires déjà bien fragilisés.

il faut plus d'une heure et demie pour rejoindre l'autoroute en toute sécurité et les lignes ferroviaires ont souvent vieilli.

que 65 millions d'euros ont été investis au cours des dix dernières années sur la ligne Aurillac-Clermont. Par ailleurs, je me suis assurée que les crédits seront bien engagés en 2018 pour garantir la pérennité de cette ligne.

Le manque de moyens n'explique pas tout ; la désorganisation de la SNCF, la perte de compétences et de savoir-faire ont des conséquences directes sur la qualité des services. Dans un contexte de mutations majeures de nos territoires, les transports et la mobilité doivent être une priorité de l'action publique, afin de répondre aux attentes de la population et des acteurs économiques. La fracture territoriale en termes de mobilité est, dans nos territoires ruraux, une réalité qui ne peut perdurer. Il ne s'agit pas d'opposer le monde rural au monde urbain, mais il n'en demeure pas moins que les métropoles ont capté l'essentiel de la croissance, tandis que des territoires se dévitalisent, malgré les efforts des élus. Le 9 décembre 2017, nous avons été contraints de bloquer les trains sur l'axe Saintes-Bordeaux. En effet, l'absence de travaux de maintenance a engendré des limitations de vitesse, induisant un allongement des temps de parcours pour les usagers et une qualité de service moindre. au soir, j'obtenais enfin un rendez-vous avec votre cabinet, madame la ministre. Je vous en remercie, mais j'attends toujours une réponse, que vous allez peut-être m'apporter aujourd'hui. Je déplore qu'il faille faire entendre fortement « nos voix sur les voies » pour être Cette baisse de performance aura des incidences sur tous les trains circulant sur l'axe Bordeaux-Saintes-Nantes, et ce, j'imagine, pendant plusieurs années. Ce qui nous inquiète, c'est le désengagement de SNCF Réseau des lignes n'appartenant pas au réseau structurant. Le gestionnaire d'infrastructures ne pourra contribuer au financement de leur renouvellement qu'à hauteur des économies de maintenance liées à ces opérations, avec une implication de l'ensemble des parties prenantes dans le cadre des contrats de plan État-région.

Mme la ministre. Monsieur le sénateur, la difficulté que vous soulignez montre, une fois de plus, la très grande fragilité de notre réseau ferré national, qui, je le redis, a souffert de décennies de sous-investissement.

Ce contrat cible les investissements sur le réseau le plus fréquenté, le traitement des lignes

les lignes ferroviaires du réseau secondaire sur la période 2015-2020. Il est clair que, avec cette enveloppe, on ne peut répondre à la totalité des besoins. En effet, l'ordre de grandeur des financements qu'il faudrait dégager pour assurer la pérennité de l'ensemble de ces lignes est de l'ordre de 5 milliards d'euros. Je connais la situation

un EPIC regroupant l'ensemble des services de mobilité et un EPIC de tête chargé d'assurer la cohérence du réseau. Je voudrais souligner que l'architecture générale découle des règles européennes, lesquelles prévoient une séparation entre le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires. Par le passé, cela avait conduit à une organisation RFF-SNCF dissociant la gestion opérationnelle de l'infrastructure

plan des préoccupations la modernisation de l'infrastructure ferroviaire. L'organisation issue de la réforme de 2014 est conforme au cadre fixé par les directives européennes. Des questions ont été soulevées, notamment sur la place des gares dans cette organisation. Cela fait partie des sujets examinés dans le cadre de la mission globale confiée à Jean-Cyril Spinetta. Des propositions avaient été faites, y compris par les parlementaires,

était privatisée et si le service de transport était totalement ouvert à la concurrence. Nous ne croyons pas à ces sornettes libérales. Il n'est plus à démontrer que toutes les expériences menées en ce sens ont conduit à une réduction du service rendu aux usagers, à une hausse des tarifs et à des problèmes de sécurité.

ce qui entraîne la suppression de certaines dessertes et l'abandon de certaines activités, comme les trains de nuit. Elles sont liées au désengagement des pouvoirs publics de ce service d'intérêt général,

Mme la ministre. Madame la sénatrice, je ne veux pas laisser penser que la nation ne consacrerait pas des sommes importantes au soutien au transport ferroviaire.

à 10 milliards d'euros, soit un ratio tout à fait comparable à ceux que l'on peut observer chez nos voisins européens. Je voudrais aussi souligner l'importance de l'engagement dans la durée que constitue le contrat entre l'État et SNCF Réseau. tend à donner une vision pluriannuelle du niveau des investissements qui doivent être réalisés sur notre réseau. À la suite de la réflexion conduite par Jean-Cyril Spinetta, des ajustements pourront être apportés, notamment sur la soutenabilité des trajectoires de péage. Il faudra également vérifier que les 3 milliards d'euros qu'il est prévu de consacrer à l'entretien et à la régénération des réseaux répondent bien aux besoins pour ramener rapidement notre réseau ferroviaire aux standards attendus au XXI siècle. En tout cas, je ne voudrais pas laisser croire qu'il n'y aurait pas de soutien public au développement du transport ferroviaire. L'ensemble du modèle économique mérite

le moins que l'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas restée inactive, et je tiens à saluer votre engagement. Au quatrième trimestre de 2017, vous avez organisé les Assises de la mobilité et lancé de grands chantiers de réflexion sur les principales infrastructures.

Néanmoins, l'ensemble des acteurs de la mobilité ont d'ores et déjà besoin de voir se dégager une ligne directrice. Tout se joue sur le rôle qui sera assigné demain à la SNCF. L'alternative est la suivante : soit la SNCF continue d'être un acteur de la mobilité parmi d'autres, principalement concentré sur la grande vitesse ; soit, au contraire, on lui assigne un objectif prioritaire d'aménagement et de désenclavement pour en faire la colonne vertébrale de la mobilité sur l'ensemble du territoire national. Là réside la question clef, parce que, dans la première hypothèse, tous les autres acteurs de la mobilité-

si la priorité est donnée à la SNCF, leur rôle sera de compléter un maillage ferroviaire développé et performant, sur lequel ils n'auront plus qu'à se greffer. Ma question est donc très simple : la SNCF constituera-t-elle demain l'axe central de l'intermodalité en France ? La parole

Toutefois, débattre de l'avenir de la SNCF, c'est en quelque sorte vouloir résoudre une équation complexe, dont l'une des principales inconnues, pour les parlementaires que nous sommes, est la contribution financière de l'État à la réduction de la dette de SNCF et au financement des projets ferroviaires régionaux. En Dordogne, plusieurs décisions sont attendues avec impatience tant par les citoyens et les usagers par les élus locaux, qui sont très fortement sollicités. C'est notamment le cas s'agissant de la ligne Libourne-Bergerac-Sarlat, qui illustre parfaitement à mes yeux cette problématique. Je vous ai interrogée à plusieurs reprises sur ce dossier, sans obtenir de réponse de votre part. C'est pourquoi je réitère ma question.

? Quelle sera la participation de l'État ? J'ose espérer que votre réponse sera aussi claire que celle que vous avez apportée à ma collègue sénatrice du Cantal, car je considère que la Dordogne est un département rural aussi enclavé

Mme la ministre. Monsieur le sénateur, nous avons déjà en effet eu à plusieurs reprises l'occasion de parler de la ligne Bergerac-Libourne, qui fait partie des nombreuses lignes régionales de Nouvelle-Aquitaine accusant un retard important en termes d'entretien.

Vous le savez, un travail est engagé au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, en lien avec l'État, pour définir les priorités d'investissement dans ce contexte. Je ne doute pas qu'il devrait conclure au caractère prioritaire de la ligne Libourne-Bergerac-Sarlat, compte tenu de sa fréquentation et de sa compétitivité par rapport aux alternatives routières. Une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés tient à la réévaluation du coût des travaux qui a été faite par SNCF Réseau postérieurement à la conclusion du contrat de plan État-région. Afin de pouvoir disposer de tous les éléments, j'ai demandé à SNCF Réseau d'avancer

Les débats des derniers mois au sein de la commission de l'aménagement du territoire ont mis au jour les inquiétudes des sénateurs quant à la place du transport régional dans le contrat de performance de la SNCF. Si lors de son audition, en avril dernier, M. Jeantet, le PDG de SNCF Réseau, semblait se féliciter que 500 millions d'euros soient affectés aux lignes régionales, alors qu'il faudrait entre 2,5 milliards et 3 milliards d'euros, il a également déclaré qu'il entendait augmenter ce budget pour atteindre le milliard d'euros au terme du contrat de performance. Plusieurs questions se posent. Ce contrat est signé pour dix ans, et il serait souhaitable de connaître le rythme annuel de progression du budget dédié au transport régional. En outre, nombreux sont les sénateurs qui se sont interrogés sur la sincérité des ambitions de ce contrat reposant sur des engagements financiers de l'État et des régions, lesquels ne sont à ce jour aucunement garantis. On peut d'autant plus être inquiet que le président de l'association Régions de France avait regretté que l'avis des régions sur le contrat n'ait pas du tout été pris en compte, alors qu'elles cofinancent largement les investissements ferroviaires locaux. des activités ferroviaires et routières, rendu le 29 mars 2017 et faisant état « d'hypothèses économiques fragiles et peu crédibles » ... Il est donc nécessaire que l'État clarifie ses intentions sur le financement du transport ferroviaire régional et sur les moyens qu'il affectera aux contrats de plan État-régions. Les régions sont, on peut le comprendre, extrêmement prudentes, et je ne voudrais pas revivre dans ma région, en matière de transport, la situation que nous connaissons aujourd'hui s'agissant du financement de la réhabilitation du logement minier : faute d'engagement de l'État, le président du conseil régional a différé, à juste titre, la mobilisation des crédits régionaux. Je rappelle aussi les enjeux, pour le département du Pas-de-Calais, en particulier pour le bassin minier, liés au Réseau express Grand Lille, qui doit relier Lille à Hénin-Beaumont, et aux investissements financiers des collectivités. Aujourd'hui, les retours sur investissements urbains ne sont pas garantis.

le sénateur, un contrat ambitieux a été signé entre l'État et SNCF Réseau pour donner de la visibilité, notamment, sur la trajectoire de régénération pour les dix prochaines années.

-que des priorités doivent être définies, région par région, quant aux lignes pouvant faire l'objet d'une régénération et d'une modernisation.

des infrastructures dont la mise à niveau est très fortement attendue par nos concitoyens. Ces contrats se poursuivent,

pour désenclaver les territoires ruraux, auxquels nous sommes très attachés ? La parole

des gares, des fréquences de desserte et de l'entretien du réseau. Nous constatons avec incompréhension l'accroissement des difficultés d'année en année. Pourtant, le train aurait pu être un formidable outil de développement et d'aménagement du territoire, ainsi que l'alternative à la voiture, que l'on nous supplie de moins utiliser. Le train s'éloigne progressivement de nos réflexes en matière de transport. Sachez, madame la ministre, que les citoyens des territoires ruraux contribuent eux aussi, par leurs impôts, au financement du déficit de la SNCF.

par un allongement des temps de parcours et par la nécessité pour les trains d'emprunter un autre itinéraire. Je suis bien consciente du désagrément causé aux voyageurs,

L'association de défense des consommateurs UFC-Que choisir vient d'interpeller les pouvoirs publics sur la dégradation de la qualité de service des trains du quotidien et sur les conditions, apparemment très inégales dans le pays, d'indemnisation des usagers victimes de retards ou d'annulations de trains.

qu'éprouvent des millions d'usagers pour aller et venir entre leur domicile et leur lieu de travail. Ces services de transport que l'on peut qualifier « de première nécessité » occupent le vingt-et-unième rang européen en matière de ponctualité et, pour diverses raisons, dont l'indispensable rénovation du réseau, connaissent une tendance préoccupante à la dégradation de la qualité de service. Pour le premier semestre de 2017, l'UFC-Que choisir fait état de 11 % de TER annulés, de 15 % d'usagers exposés à des retards aux heures de pointe, et relève que seule une ligne sur les treize que compte le Transilien en région parisienne remplit ses objectifs contractuels de ponctualité. Elle impute 59 % des retards constatés à la gestion des circulations par SNCF Mobilités, indépendamment de tout incident imputable à l'infrastructure ou aux travaux Alors que la SNCF a mis en place un système d'indemnisation des retards et annulations de trains souvent considéré comme excessivement procédurier ou décourageant, on apprend que deux tiers des régions n'ont pas mis en place un tel dispositif

Je vous serais reconnaissant, madame la ministre, de bien vouloir faire toute la lumière sur cette curiosité nationale qui voudrait que les droits des clients des trains commerciaux de la SNCF soient

pour les trains qui relèvent de sa responsabilité ; il appartient aux autorités organisatrices, dans le transport ferroviaire comme dans le transport urbain, de définir des régimes de pénalités applicables à leurs opérateurs et des régimes d'indemnisation applicables à leurs voyageurs. La négociation des prochains contrats par les autorités organisatrices sera peut-être l'occasion de préciser ces points,

Il a également été reconnu comme étant le sixième meilleur réseau ferroviaire du monde. Malgré cela, nous constatons régulièrement de nombreux défauts. Je ne reviendrai pas sur les diverses perturbations que de nombreux Français ont subies au cours du mois de décembre, et qui ne font malheureusement qu'aggraver leur mauvaise opinion des services de la SNCF.

Il serait en effet opportun d'ouvrir aux régions qui le souhaitent la possibilité de participer à ce financement. Y êtes-vous favorable, madame la ministre ? Je profite de ce court temps de parole pour vous interroger sur votre engagement à l'égard su projet franco-suisse du RER Sud-Léman. La ligne ferroviaire d'Évian-les-Bains à Saint-Gingolph est le dernier maillon de la boucle ferroviaire du lac Léman. Vous connaissez notre combat pour le désenclavement du territoire du Chablais : ce projet de réouverture aux voyageurs- j'insiste sur ce point - de la ligne Sud-Léman permettra de désenclaver l'est du Chablais. SNCF Réseau a donné son feu vert, les collectivités françaises ainsi que les cantons suisses de Vaud, du Valais et de Genève sont également favorables au projet, et la région vient de reconfirmer son engagement. Considérant l'importance de ce projet pour notre territoire, la réaffirmation des soutiens côté français est un bon signal envoyé à nos voisins Suisses, à l'heure où ils fixent leurs priorités en matière de financement du ferroviaire à l'horizon 2035 : le RER Sud-Léman pourrait bénéficier de fonds de la Confédération helvétique. En tant que président du comité de pilotage du projet du RER Sud-Léman, je me permets de vous demander, madame la ministre, d'affirmer le soutien du Gouvernement français. La parole est à Mme la ministre.

réunirai, le 15 février prochain, le comité ministériel sur la sécurité ferroviaire et sur la sécurité aux passages à niveau pour réaffirmer l'engagement de l'État.

socialiste et républicain. À l'automne, le Président de la République a annoncé son souhait de réformer drastiquement le régime spécial de retraite des cheminots, en contrepartie d'un allégement partiel

de l'État. Si elle pouvait l'être, cela permettrait de financer de nouvelles infrastructures, comme nous le souhaiterions, et surtout de viabiliser un groupe dont l'actif net est virtuellement inexistant

d'agrégation de mobilités, ou bien n'est-ce qu'un moyen d'embellir à peu de frais la corbeille de la mariée en vue d'une vente à la découpe de la SNCF qui ne dit pas son nom, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des lignes TER et TGV d'ici à décembre 2019 et à janvier 2021 ? Madame la ministre, j'ai apprécié l'exercice des Assises de la mobilité, auxquelles j'ai pris part. Je vous ai entendu, lors de la conclusion de ces assises, annoncer

d'aborder ce sujet avec sérénité, dans la concertation, pour que l'ouverture à la concurrence se fasse au bénéfice des régions et des voyageurs, tout en rassurant les cheminots sur leur avenir. La parole est à M. Jean Sol, pour

Je ne peux m'empêcher de penser, en cet instant, aux familles meurtries par ce drame et au maire de Saint-Féliu-d'Avall, Robert Taillant, dont l'exemplarité face à cette tragédie est à souligner.

Si je suis, comme vous et de nombreux élus, conscient de l'impérieuse nécessité de pouvoir bénéficier d'un nouveau dispositif de programmation des investissements pour les transports de demain, je considère que celui-ci doit se bâtir sur la base du respect de l'égalité de nos concitoyens face à la mobilité et de la correction des inégalités entre territoires. Force est de constater que Perpignan fait encore partie, malheureusement, des villes situées à plus de cinq heures de la capitale. Force est de constater que les lignes à grande vitesse traversent la France des régions, mais s'arrêtent aux portes de Montpellier, alors que l'Espagne a inauguré une LGV Madrid-Barcelone-Figueras. Force est de constater le manque d'investissements de l'État

transformation urbaine de nos villes, du tourisme, de l'économie et de la compétitivité de nos territoires. En termes sociétaux, la multiplication des camions sur les routes est devenue l'un des premiers facteurs d'insécurité routière et de pollution atmosphérique. Comment nier, en ce XXI siècle, la nécessité de finaliser enfin ce projet, attendu depuis plus de trente ans par des usagers aujourd'hui excédés et prêts à se mobiliser au côté des élus que nous sommes

Bien que la France constitue la proue de l'Europe sur l'Atlantique, le port du Havre ne figure pas dans les cinquante premiers ports mondiaux, et plus de 50 % des marchandises arrivant en France transitent par des ports étrangers. Or, en matière de transport de marchandises, les enjeux maritimes, fluviaux et ferroviaires se rejoignent. Pendant ce temps, après avoir repris et modernisé les ports du Pirée, en Grèce, la Chine ambitionne de contrôler le réseau ferroviaire de ce pays pour mieux irriguer le coeur de l'Europe, et, avant même la montée en puissance de l'ambitieux projet de la route de la soie,

l'on vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour l'autoroute ferroviaire atlantique. Je pense que le ferroviaire doit reprendre toute sa place dans le transport de marchandises ; cela passera par des choix en matière d'infrastructures dont le Conseil d'orientation des infrastructures est

d'une très grande difficulté de maîtrise technique par notre entreprise publique. Au-delà, c'est la situation globale du groupe qui me paraît préoccupante. La dette, qui atteint désormais qui atteint désormais plus de 50 milliards d'euros selon le rapport de l'Agence des participations de l'État, avec une projection à 60 milliards d'euros à

passer par un assainissement financier de SNCF Réseau et par l'ouverture à la concurrence pour stimuler SNCF Mobilités, afin d'améliorer sa compétitivité et de rendre un meilleur service aux usagers. J'aimerais, madame la ministre, connaître votre position sur ces sujets.

d'aborder simultanément tous les sujets : l'état de l'infrastructure- c'est notamment l'objet des travaux réalisés dans le cadre du Conseil d'orientation des infrastructures, auquel vous participez -, le modèle économique,

dans un contexte où l'augmentation de la fréquence des dessertes vers la gare du Nord n'est plus possible aux heures de pointe ; j'ai quinze ans d'expérience quotidienne de ce trajet

entre la ligne Creil-Paris-Nord et l'aéroport de Roissy, ainsi qu'en l'aménagement de gares à Roissy, à Survilliers, à Chantilly et à Amiens. Compte tenu des enjeux, le conseil départemental de l'Oise, sous la présidence de notre collègue Édouard Courtial et en lien avec le président Xavier Bertrand, a pris l'initiative de réunir les financements de toutes les collectivités locales concernées. Ma question est simple, madame la ministre : quand comptez-vous donner une suite favorable à ce projet, qui ne saurait avancer à un train de sénateur ?

Il s'agit d'un nouvel outil de gestion des compétences et des parcours professionnels à la main des partenaires sociaux et dont se sont saisies dans le Nord deux entreprises, PSA et Pimkie, la presse s'en étant largement fait l'écho ces derniers jours.

l'accord doit être homologué par l'administration, qui contrôle ensuite son application. Elle s'assurera notamment qu'il ne s'agit pas de préretraites déguisées et que l'accord prévoit des mesures d'accompagnement et de reclassement. En troisième lieu, les salariés doivent être volontaires pour bénéficier des mesures négociées par les partenaires sociaux. L'accord de RCC permet aux salariés de bénéficier, en plus des indemnités de chômage, de toutes les mesures ayant été négociées, par exemple des indemnités spécifiques ou des mesures de reclassement et d'accompagnement. De surcroît, ces indemnités relèvent d'un régime social et fiscal favorable, comme dans le cas des plans de départs volontaires. Il apparaît donc qu'il s'agit d'un outil permettant de ménager le climat social dans l'entreprise, car plus consensuel et plus sûr sur le plan juridique qu'un plan

de téléphonie mobile est une attente majeure de nos concitoyens, en particulier de ceux qui vivent en zone rurale et entendent bien des promesses depuis longtemps. Il s'agit d'un enjeu primordial en matière d'aménagement des territoires, et le Président de la République s'est engagé à généraliser une couverture mobile de qualité avant 2020. Aux côtés de M. Jacques Mézard, vous avez annoncé, dimanche soir, avoir abouti à un accord avec les opérateurs de télécommunication, accord qui prévoit un investissement de plus de 3 milliards d'euros supplémentaires au titre de cet engagement. Il s'agit d'une mesure de justice indispensable à la cohésion de notre pays et surtout à l'égalité des territoires. Toutefois, je vous rappelle que de telles promesses ont déjà été faites,

quelles simplifications administratives allez-vous mettre en oeuvre ? Enfin, il me paraît important que vous nous indiquiez comment vous vous êtes assuré que cet accord était, du point de vue de l'État, un bon accord et quel sera le rôle des élus locaux, qui sont aujourd'hui découragés, parce qu'ils n'ont aucune prise sur les décisions des opérateurs. La

Ils pourront prochainement mettre en ligne leurs dossiers, qui seront examinés par les universités en fonction d'attendus que celles-ci élaborent en ce moment. Au travers de ces attendus, en dehors de tout cadre légal, plusieurs universités demandent aux candidats et candidates des lettres de motivation, des justificatifs de stage ou encore des diplômes comme le Elles ont parfaitement compris le sens de votre projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants et mettent en place une sélection drastique que vous n'assumez pas politiquement. Tout se passe donc comme si les dispositions de votre projet de loi étaient appliquées avant même d'avoir été discutées par la Haute Assemblée, qui en débattra les 7 et 8 février prochains.

républicain citoyen et écologiste se réserve la possibilité de déférer devant les juridictions administratives les actes des universités qui seraient contraires aux dispositions du code de l'éducation tel qu'il s'applique aujourd'hui.

Personne ne sera laissé au bord du chemin : les dispositions nécessaires ont été prises pour que ce mécanisme d'information et d'orientation permette de traiter l'ensemble des demandes.

pour 80 % des contribuables français, ceux dont le revenu est inférieur à 2 500 euros par mois. Cette mesure est parfaitement financée. La trajectoire budgétaire est respectée. Nous avons même réussi à obtenir une amélioration du déficit budgétaire de 6 milliards d'euros en 2017, preuve que les comptes publics de la France sont bien tenus sous le gouvernement d'Édouard Philippe ! Il nous reste à trouver non pas 19 milliards d'euros, mais 8,5 milliards d'euros pour financer la suppression totale de la taxe d'habitation. Trois pistes sont sur la table

et je salue le fait que la France y ait été particulièrement bien représentée, par plus de 320 start-up, soit la deuxième délégation après celle des États-Unis.

et ses territoires ont des atouts incroyables pour faire rayonner la « » dans le monde. Nous demeurons une grande nation d'innovation et de créativité Cependant, les chiffres du commerce extérieur publiés la semaine dernière par les services des douanes font état d'un déficit abyssal de 60 milliards d'euros sur douze mois, à nuancer ces succès. Oui, nous innovons. Oui, nous sommes créatifs. Oui, notre écosystème de start-up est dense et performant, mais il peine à mettre en oeuvre une véritable stratégie de reconquête de parts de marchés à l'étranger. Notre compétitivité au sein même de l'Union européenne ne cesse de s'éroder. À titre de comparaison, l'Allemagne affiche, elle, un excédent commercial de 227 milliards d'euros entre janvier et novembre 2017. Nos PME innovantes exportent peu, n'ont souvent pas la taille critique pour s'attaquer aux marchés étrangers et ont du mal à trouver les financements nécessaires à leur croissance. Monsieur le ministre, ma question est simple quelle est votre stratégie pour faire en sorte que la « » soit davantage qu'une opération de communication à l'étranger et devienne une réalité industrielle qui place la France aux premiers rangs mondiaux de l'économie de demain ?

De manière plus large, personne ne peut se résigner à voir se creuser, depuis le début des années 2000, le déficit commercial extérieur de la France. Ce dernier est le reflet de la perte de compétitivité de notre économie. Certes, nous innovons, monsieur le sénateur,

d'investir et d'innover. Le Fonds pour l'innovation de rupture, que nous allons mettre en place dès ce mois-ci avec 10 milliards d'euros de dotation, aura pour objet de financer l'innovation de rupture, laquelle nous permettra de continuer à être une nation conquérante sur les marchés extérieurs. Personne ici,

réforme ne consiste pas en une simple suppression ; il s'agit d'un dégrèvement, l'État se substituant donc au contribuable local. Cependant, l'histoire budgétaire nous rappelle que toute compensation reste fragile.

nombreux élus craignent- à raison, l'histoire ayant laissé des traces -que ce dégrèvement ne remette en cause l'autonomie financière des communes, qui est pourtant un principe constitutionnel. L'État manquant lui-même de ressources, il est étrange qu'il se permette de priver des leurs les collectivités, étranglées financièrement depuis plusieurs années. Le Conseil constitutionnel a validé la loi de finances, mais il a émis de sérieuses réserves concernant ce dégrèvement, qui portera dans un futur très proche des atteintes graves au principe constitutionnel de libre administration des collectivités. La réponse apportée par M. le ministre de l'économie et des

! Personne ne peut se satisfaire de la complexité de la fiscalité locale actuelle. Si vous vous satisfaites de la taxe d'habitation,

! C'est l'honneur de cette majorité que d'avoir le courage de réformer en profondeur la fiscalité locale. C'est l'honneur de cette majorité que de répondre aux attentes de nos concitoyens. C'est l'honneur de cette majorité que de rendre en moyenne 200 euros de pouvoir d'achat en 2018 à 80 % des contribuables, les plus modestes, par la suppression de la taxe d'habitation. Vous la supprimez

des inquiétudes fortes demeurent, car il ne s'agit que d'une étape du long processus législatif européen. Pour que cette avancée acquière force de loi, elle doit être validée européen. La pêche électrique consiste à envoyer un courant électrique dans des électrodes placées sur les filets, afin de paralyser les poissons et ainsi de les capturer plus facilement. Ce procédé redoutable et cruel était déjà interdit depuis 1998, mais les Pays-Bas, notamment, profitaient d'une dérogation accordée à titre exceptionnel pour une quinzaine de navires. Nos pêcheurs français, qui refusaient d'y avoir recours, en subissaient les conséquences en termes de ressource, la mer du Nord devenant bel et bien un cimetière marin. Alors même que nos pêcheurs modernisent depuis plusieurs années leur flotte et leurs techniques, afin d'offrir aux consommateurs des produits de qualité issus d'une pêche responsable et durable, leurs efforts sont compromis par un contexte juridique et politique

Le Gouvernement s'engage-t-il à faire preuve de la même vigilance dans les eaux de l'océan Indien, pour que ces méthodes ravageuses ne s'y implantent pas ? De fait, il y a bel et bien un déplacement des flottes vers les mers de l'hémisphère sud, encore poissonneuses.

L'année 2017 a de nouveau révélé la vétusté du parc ferroviaire français, alors que le train est le premier moyen de transport collectif à distance. Nos concitoyens ont en effet été victimes

la section Libourne-Bergerac, que vous venez d'évoquer, fait partie des nombreuses lignes régionales qui souffrent d'un défaut d'entretien et d'investissement depuis des années. Vous le savez, alors qu'au cours des dix-huit derniers mois nous avons inauguré quatre lignes à grande vitesse, ce sont plus de 5 300 kilomètres de réseau qui font l'objet de ralentissements du fait de ce sous-entretien et de ce sous-investissement. C'est dans ce contexte que le Gouvernement a donné la priorité à l'entretien et à la modernisation des réseaux. Je ne me risquerai pas à vous dire que nous allons remédier en quelques mois à des décennies de sous-entretien et de sous-investissement, en 2018, ce sont 5,2 milliards d'euros qui vont être consacrés par SNCF Réseau à cette priorité. Par ailleurs, il est prévu d'allouer 1,5 milliard d'euros aux lignes secondaires dans le cadre des contrats de plan État-régions. Pour autant, ces ressources ne permettront pas de traiter l'ensemble des lignes qui connaissent aujourd'hui des difficultés. C'est pourquoi un travail spécifique est engagé au sein de la région Nouvelle-Aquitaine.

Libourne-Bergerac, sera retenue parmi les lignes prioritaires, compte tenu de son trafic et de sa compétitivité par rapport aux alternatives routières. Il nous Il nous faudra aussi optimiser le programme de travaux, aujourd'hui évalué à 90 millions d'euros. C'est le sens des études engagées depuis la fin de l'année 2017 pour cibler au mieux les travaux sur cette ligne. état de cause, vous pouvez compter sur ma détermination à trouver des solutions pour ces petites lignes ferroviaires en difficulté.

Les principales associations locales d'aide aux migrants ont annoncé qu'elles boycotteraient la rencontre avec le Président de la République prévue ce mardi, lui reprochant un manque d'écoute et de dialogue. Derrière cette opération de communication du Président de la République, derrière cette volonté gouvernementale de lutter contre l'immigration économique et de rendre plus efficaces les expulsions des déboutés du droit d'asile,

La France est un grand pays qui doit faire face à ses responsabilités, mais elle ne saurait évidemment y parvenir seule. L'erreur initiale a été d'avoir laissé s'installer à Calais de 7 000 à 8 000 personnes dans des conditions d'hygiène, de sécurité et d'abandon épouvantables. qui avait été mis en place, sous le précédent quinquennat, dans le centre d'accueil Jules-Ferry, était à la fois professionnel et surveillé et n'avait donné lieu à aucun accident. Aujourd'hui, il n'est plus question de réinstaller quoi que ce soit à cet endroit, mais d'aménager un lieu dédié, où des migrants puissent être secourus et accueillis dans des conditions dignes d'un grand pays moderne. C'est une exigence républicaine. Il est tout aussi indispensable d'obtenir des autorités britanniques qu'elles prennent désormais leur part du problème. À Calais, la population attend du Gouvernement des réponses quant à ses propres difficultés d'emploi,

Madame Van Heghe, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, se trouve naturellement aux côtés du Président de la République à Calais. Cette visite a pour but de rencontrer tous ceux qui travaillent sur le thème de la politique migratoire : élus, associations et forces de sécurité.

que d'accueillir celles et ceux qui fuient les théâtres de guerre, celles et ceux qui, dans leur pays, sont victimes de persécutions pour des raisons politiques, ethniques ou religieuses. L'accueil inconditionnel des migrants est respecté dans notre pays. ensuite, car on ne saurait garantir le droit d'asile sans maîtriser les flux migratoires ni reconduire à la frontière ceux

appel au secours, celui des enseignants du lycée Joseph-Gallieni de Toulouse, qui accueille 1 000 élèves, du CAP au bac professionnel et technologique. Mardi dernier, les enseignants de cet établissement étaient en grève pour dénoncer une situation inouïe, qui dure depuis des années et qui ne cesse d'empirer 150 élèves « très difficiles », parfois délinquants, font régner la terreur dans ce lycée. Ils y ont pris le pouvoir : agressions verbales, menaces, coups, jets de pierres et de canettes à l'encontre du personnel de l'établissement humiliations des élèves les plus faibles ; exclusions des filles de certains espaces de convivialité ; vols ; généralisation des bagarres, toujours plus violentes ; déclenchements d'incendies ... Tout cela, bien sûr, sur fond de trafic de drogue. Les surveillants de l'établissement sont aujourd'hui dépassés, épuisés. Les professeurs confient venir travailler la peur au ventre- on les comprend

L'accueil d'élèves particulièrement difficiles conduit à remettre en cause les chances de réussite de tous ceux qui, dans ces établissements, souhaitent travailler. ne croyez-vous pas qu'il est temps de prendre à bras-le-corps ce dossier et de se poser la question de la création d'établissements d'accueil adaptés à ces situations ? Ne croyez-vous pas qu'il convient de repenser en profondeur l'organisation des parcours scolaires

dès la semaine dernière, l'équipe de direction pour envisager, avec les autorités des collectivités locales, les moyens d'aménagement nécessaires pour cet établissement. L'inspecteur d'académie et les services du rectorat recevront ce soir

Comme M. Gay, je voudrais revenir sur le lancement de la plateforme d'inscription dans l'enseignement supérieur, dite « Parcoursup », présentée lundi à grand renfort de relais médiatiques, d'échanges et même d'un déjeuner avec des lycéens. Certes, l'ancienne procédure admission post-bac a connu des dysfonctionnements importants et tout le monde s'accorde ici sur l'absolue nécessité d'éviter le recours au tirage au sort pour les admissions dans les filières dites « sous tension

Aucun débat de fond ne peut réellement s'instaurer. C'est un déni de démocratie assez scandaleux, qui en dit long sur votre considération du Parlement. Pourquoi nous faire voter une loi que vous avez en réalité déjà mise en application ? Comment justifiez-vous que toute modification significative du texte par le Sénat soit systématiquement rejetée ?

pense qu'il était urgent d'agir. Je ne doute pas que nous puissions nous retrouver, ensemble, pour débattre de ce texte, l'améliorer et faire en sorte qu'il entre en vigueur dans les meilleures conditions,

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur l'état du service public dans les transports en région Île-de-France, organisé à la demande du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les Franciliennes et les Franciliens qui empruntent les transports en commun ne supportent plus la galère qu'elles ou ils vivent au quotidien : retards, annulations, incidents divers, inconfort générant stress et fatigue ... Cette exaspération légitime nourrit un sentiment de déclassement et d'abandon que nous ne pouvons ignorer. Quant aux personnels de la RATP et de la SNCF, dont il faut saluer l'engagement professionnel, ils sont en souffrance face à la dégradation de leurs conditions de travail. Si la question du service public des transports et de sa dégradation se pose sur l'ensemble du territoire national, comme nous l'avons vu lors du débat précédent, les caractéristiques de la région capitale en font une question spécifique sur cet espace qui concentre 5 millions de voyageuses et de voyageurs par jour. Parler transports, c'est aborder la question de l'aménagement. Le droit à la mobilité ne peut se penser en dehors du droit au logement accessible ni des problématiques d'accès à l'emploi et aux services publics. Tenir ces quatre exigences, c'est permettre un aménagement équilibré et une meilleure qualité de vie pour les Franciliennes et les Franciliens. Or nous avons hérité, depuis des décennies, d'un déséquilibre entre l'est et l'ouest régional. Pour faire vite, les bureaux sont à l'ouest et les logements à l'est, ce qui entraîne des mouvements de transports trop importants. Le développement urbain a également créé de nouveaux besoins de mobilité encore sans réponse aujourd'hui. Un rééquilibrage entre bureau et logement et une réelle réflexion sur l'étalement urbain constituent donc un premier élément de réponse aux problèmes de transport. si l'enjeu des transports collectifs est un enjeu majeur, c'est aussi parce qu'il touche à des défis environnementaux et sanitaires. Trop de camions et de voitures saturent le réseau. Je rappelle que nous déplorons 6 000 morts par an en Île-de-France du fait de la pollution- sans compter les coûts induits estimés, à l'échelle de la France, à 101 milliards d'euros par an. Il est donc urgent d'inverser la tendance en engageant un report modal de la route vers le rail et vers le fluvial, pour les voyageurs comme pour les marchandises.

Respecter les engagements liés à l'accord de Paris pris dans le cadre de la COP21 doit donc nous conduire à adopter des politiques qui favorisent le rail face à la route, le collectif face à l'individuel. Grande question de santé publique, l'accessibilité des transports en commun constitue également un enjeu social. Trop de nos concitoyennes et de nos concitoyens subissent en effet une discrimination à l'embauche selon l'endroit où elles et ils résident. Et ces mauvaises conditions de transport, comme la saturation des réseaux routiers, sont un frein évident à la compétitivité des entreprises, qui ont intérêt à disposer de bonnes conditions de mobilité pour leurs salariés comme pour leur clientèle. Depuis plus de dix ans, les politiques publiques en matière de transport tiennent en un mot le désengagement de l'État. On peut même se demander si ces conditions n'ont pas été créées pour aboutir à cette situation dégradée, afin de justifier des politiques de libéralisation et de privatisation. Comment laisser entendre que l'ouverture à la concurrence pourrait être la solution aux dysfonctionnements actuels, puisque tout recul de la puissance publique entraînera un recul de l'égalité et des droits ? En effet, la mise en concurrence ne peut qu'aboutir au délaissement de la partie du territoire jugée la moins rentable- je pense notamment à la grande couronne. À la concurrence, nous préférons la complémentarité entre les différents modes de transports- le ferroviaire, le bus, les vélos -, afin d'offrir une offre cohérente et maillée sur l'ensemble du territoire, ce qui implique, mais j'y reviendrai, un renforcement de la maîtrise publique de ce secteur. L'ouverture à la concurrence, c'est également le social, économique et environnemental et des prises de risque pour la sécurité des usagers et des personnels. Nous pensons donc qu'il faut en finir avec cette logique libérale en transformant et en améliorant le service public des transports collectifs. Cela suppose notamment d'abandonner les projets qui ne répondent pas aux besoins des Franciliennes et des Franciliens. Je pense ici au projet privé CDG Express, qui ne vise qu'à satisfaire les usagers d'affaires qui pourront dépenser 24 euros pour aller de l'aéroport à Paris. Ce projet, qui bénéficie d'un fort soutien public-

de même du prolongement de la ligne 14. Je ne pense pas qu'un seul sénateur ici présent soit satisfait des conditions de transports dans la région Île-de-France. Je ne crois pas davantage que notre groupe soit le seul à remarquer un déséquilibre entre l'est et l'ouest, avec une concentration d'entreprises autour de La Défense. Si le constat est largement partagé, la question qui nous est posée, mes chers collègues, est celle des actions que nous sommes prêts à engager pour remédier à cette situation. Or les choix politiques faits depuis des dizaines d'années ne permettent pas de développer un réseau de transports publics digne du XXI siècle.

participant à la nécessaire transition écologique, il faut, au contraire, améliorer et renforcer le service public des transports. Pour ce faire, il convient de s'engager dès à présent dans des travaux visant à rénover et faire évoluer le réseau francilien existant. Nous avons besoin d'investissements massifs pour mener à bien les chantiers programmés, mais aussi pour assurer une maintenance de qualité ou renouveler le matériel roulant, même si nombre d'efforts ont été faits de ce point de vue sous la précédente mandature régionale. Ainsi, il est urgent d'investir massivement sur l'ensemble des lignes du RER, véritable point noir du réseau régional, et de poursuivre le développement et le maillage des réseaux de bus. Il est urgent que les opérateurs publics que sont la SNCF et la RATP développent une politique d'embauche, afin d'améliorer les services aux voyageurs. Concernant le fret, les triages et les infrastructures doivent retrouver une pleine activité, et les emprises foncières être préservées. Pour tous ces investissements, notre sensibilité politique formule, aux niveaux local et national, d'autres pistes de financement nourries par le dialogue avec les syndicalistes, les usagers et les élus.

grâce à la mobilisation que nous avons contribué à impulser. Je l'ai vécue en tant que conseillère régionale et administratrice du STIF, aujourd'hui Île-de-France Mobilités. Nous avons également contribué à la prise en compte, au travers de la tarification sociale, des difficultés des plus fragiles les jeunes, les privés d'emploi et les retraités. Néanmoins, aujourd'hui, la nouvelle majorité de droite remet en cause tous ces acquis, n'ayant de cesse, notamment, d'augmenter le prix du pass Navigo. Pourtant, les départements du Val-de-Marne et de Paris viennent d'adopter des mesures de tarification spéciale et de gratuité en faveur des retraités.

matière. Je pense non seulement aux usagers, mais aussi au personnel. Madame la ministre, les usagers, les associations, les comités de ligne et les syndicats attendent, avec nous, des réponses extrêmement précises aux propositions que nous formulons et qui sont largement partagées. En réalité, l'apport de notre

à la fois pour mettre un coup d'arrêt aux galères vécues par les Franciliennes et les Franciliens dans les transports en commun et pour redonner au fret ferroviaire la place qui doit être la sienne dans l'intérêt de toutes et tous. La parole

Vous le savez, je suis également, de par mes précédentes fonctions, sensible aux enjeux des transports publics en Île-de-France et, plus largement, à l'offre de mobilités dans Je ne reviendrai pas sur les sujets que nous avons pu aborder lors de notre premier débat et qui concernaient aussi l'Île-de-France. Cependant, je le constate tout autant que vous, tout ne fonctionne pas au mieux. tous la spécificité du contexte francilien et la saturation réelle des réseaux, structurés historiquement en radiale entre Paris et ses territoires limitrophes. Bien sûr, je ne m'en satisfais pas, et l'État, même s'il n'est pas autorité organisatrice des transports en Île-de-France, s'engage fortement dans la région capitale. En effet, le Gouvernement a pleinement conscience des enjeux, notamment de l'urgence de la rénovation de l'existant et de l'amélioration des conditions de transport au quotidien. également pleinement engagé pour accompagner des projets de dimension internationale à moyen terme - je pense aux jeux Olympiques de 2024 ou encore à l'organisation de la Coupe du monde de rugby en 2023 -, destinés à soutenir le développement et l'attractivité de la région capitale.

en permettant aux autorités organisatrices d'assurer le développement d'une offre de mobilités de qualité. Deuxièmement, il est nécessaire de lutter contre la pollution de l'air et d'aider les collectivités à mettre en oeuvre la transition énergétique,

les jours, mesdames, messieurs les sénateurs, l'État s'engage aux côtés des collectivités franciliennes pour l'amélioration des transports du quotidien, qu'il s'agisse du RER, du métro, du tramway ou du bus à haut niveau de service.

Pour l'année 2018, des projets prioritaires, tels que le prolongement de la ligne 11, le tram-train Massy-Évry ou encore le T9 bénéficieront de crédits de l'État. Par ailleurs, je tiens à rappeler que la RATP et la SNCF déploieront 1,6 milliard d'euros pour la régénération de leur réseau en 2018.

Vous le savez, la fin des études et l'entrée en phase opérationnelle - je pense en particulier à la ligne 15 Sud -ont conduit à préciser la réalité des coûts et des délais. Je le dis très clairement, le calendrier présenté jusqu'à présent était, pour partie, trop ambitieux. Dans ce contexte, et sans remettre en cause le projet, le Gouvernement a lancé une réflexion, confiée au préfet d'Île-de-France, sur le rythme de réalisation du projet et ses modalités de financement.

Avec la présidente d'Île-de-France Mobilités, nous avons réuni vendredi dernier les présidents de la SNCF, de la RATP et de la Société du Grand Paris, afin de leur demander de mieux se coordonner et de mieux informer sur les opérations de travaux de rénovation ou d'interconnexion en cours. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous le constatez avec moi : bien qu'il ne soit pas autorité organisatrice des transports, l'État s'engage pour l'Île-de-France et son service public de transport. Enfin, au-delà des grands projets et de la rénovation des réseaux, mon devoir en tant que ministre est aussi de permettre aux autorités organisatrices, au premier rang desquelles figure Île-de-France Mobilités, et aux collectivités comme la Ville de Paris, la région Île-de-France ou la métropole du Grand Paris de se projeter dans les mobilités du XXI siècle. Je l'ai dit tout à l'heure, tel est l'objet de loi d'orientation des mobilités qui sera présentée au printemps. C'est pourquoi, en complément de ce que l'on appelle le, la loi d'orientation des mobilités doit permettre d'offrir un cadre réglementaire incitant à aller vers plus d'innovations dans les mobilités-

la mobilité des biens et des personnes est un enjeu majeur, à la fois économique, social et environnemental. Nous devons nous assurer que nous apportons des solutions de mobilité durables à tous les citoyens, dans tous les territoires.

Mes chers collègues, je suis heureuse de saluer en votre nom la présence, dans notre tribune d'honneur, d'une délégation du Sénat pakistanais, conduite par le général Abdul Qayyum, qui effectue une mission en vue de développer nos coopérations bilatérales, en particulier dans les domaines de la défense et de l'économie. La délégation est accompagnée par notre collègue Pascal Allizard, président du groupe d'amitié France-Pakistan. Cette visite s'inscrit dans le prolongement d'un échange interparlementaire particulièrement dense et dynamique, avec la visite récente au Pakistan de délégations des groupes d'amitié de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais aussi de notre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. La richesse de cette relation interparlementaire nous rappelle que les vertus du bicamérisme vont bien au-delà de la seule fonction législative. Lors de son séjour, la délégation s'entretiendra en particulier avec notre collègue Christian Cambon, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, et effectuera plusieurs visites à caractère économique. Nous souhaitons à nos collègues pakistanais un fructueux séjour, en formant le voeu que cette session de travail interparlementaire contribue à l'approfondissement de nos coopérations et à l'éclosion, autour de valeurs partagées, d'opportunités réciproques. Nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue au Sénat français !

alors que les transports devraient être des facilitateurs du quotidien, ils sont aujourd'hui une véritable plaie dans la vie de millions de Franciliens ; du fait du manque d'investissements affectant de nombreuses lignes de notre réseau, ils sont source de difficultés réelles pour leur santé, leur emploi ou leur vie familiale.

stress, perte d'emploi ou fatigue chronique. Pourtant, les transports collectifs sont une réponse économique, sociale et environnementale viable. Personne n'a intérêt à ce que des dizaines de milliers de Franciliens s'en détournent pour prendre des transports individuels, notamment la voiture, même partagée.

? Les usagers du RER B attendent avec impatience, depuis des décennies, le doublement du tunnel du Châtelet ou le rehaussement des ponts de la partie sud, qui permettrait de fluidifier le trafic grâce à des rames à double étage. Ma question sera simple, franche et directe, madame la ministre

auxquels s'ajoutent 2,5 milliards d'euros apportés par la Société du Grand Paris sur la période 2017-2020. Tout cela permettra un programme d'investissements de 7,5 milliards d'euros sur la période du contrat de plan, auxquels s'ajoute 1,6 milliard d'euros

Mme la ministre. Monsieur le sénateur, je veux vous rassurer s'agissant de l'importance, pour le Gouvernement, du projet du Grand Paris Express. Je l'ai dit, le développement des réseaux en Île-de-France s'est fait de façon radiale,

Au moins 267 000 personnes ont été victimes d'atteintes sexuelles dans les transports en commun de 2014 à 2015. Malheureusement, ces chiffres n'auront certainement pas diminué depuis lors ! Qui plus est, c'est une fourchette basse. Sans surprise, les femmes représentent l'écrasante majorité des victimes d'agressions. Les deux tiers des victimes d'injures et d'insultes sont des femmes, tout comme la majorité des victimes de violences sexuelles. Ainsi, six femmes sur dix craignent une agression ou un vol dans les transports franciliens, contre trois hommes sur dix. Si l'anonymat des transports en commun favorise les comportements des agresseurs, c'est surtout

est également d'accompagner les opérateurs pour qu'ils puissent développer des solutions de vidéo intelligentes, afin de mieux exploiter les images de ces caméras, au profit de la sécurité des voyageurs. Nous avons enfin des systèmes d'alerte. Vous le savez, la RATP et la SNCF partagent un numéro commun, le 3117 ou le 31117, qui permet d'alerter en cas d'incivilité ou de

minutes pour un trajet direct, un mode de déplacement idéal lorsque l'on sait que le même trajet en voiture prend dans le meilleur des cas une heure, et je ne vous parle pas du pire, sachant que la moyenne quotidienne tourne autour d'une heure et demie ! Malheureusement, en Île-de-France, et plus particulièrement en Seine-et-Marne, le premier de ses départements par la taille, mais également par la croissance démographique, les déplacements relèvent de l'exploit tant les perturbations en tous genres font des transports collectifs un mode de déplacement peu fiable. La multiplication des problèmes survenus à la fin de l'année 2017 révèle trente années de sous-investissements dans les infrastructures de la SNCF, avec pour conséquence une situation qui ne pourra que se dégrader si, comme l'a réclamé Valérie Pécresse, présidente de la région, un plan ORSEC pour les transports franciliens n'est pas déclenché. En Seine-et-Marne, la voiture demeure le premier mode de déplacement. Comment demander aux Seine-et-Marnais de moins utiliser leur véhicule et, dans le même temps, les priver de transports en commun de qualité ? La ligne P est le symbole de l'abandon de la Seine-et-Marne. Cette ligne encore non électrifiée cumule les problèmes depuis de nombreuses années : insécurité, manque de personnel, matériel vieillissant et progression du nombre Pour compléter une réalité inacceptable, l'État refuse de financer les interconnexions et décide de retarder la création de la ligne 17 du Grand Paris Express, vitale pour 420 000 habitants Madame la ministre, en ce début d'année, les Seine-et-Marnais aimeraient beaucoup recevoir de votre part un signe fort. Alors que les Assises de la mobilité viennent de s'achever

de sous-investissement et de sous-entretien pendant des décennies. C'est sûr ! Nous serons ainsi conduits à réorienter fortement nos priorités en faveur des transports du quotidien, de l'entretien et de la modernisation des réseaux. Nous serons aussi amenés à faire des choix

revenir -, un département comme la Seine-et-Marne a besoin non seulement d'infrastructures lourdes, mais aussi de nouvelles solutions de mobilité, de covoiturage, d'autopartage, de transport à la demande. Je sais que la présidente d'Île-de-France Mobilités

qui traverse l'Essonne. Nous concevons les transports de demain comme il y a trente ans, alors que des projets plus adaptés aux bassins de vie, plus efficaces et moins coûteux, mais aussi plus rapides à créer- c'est très important -permettraient d'apporter des réponses à l'urgence des usagers au quotidien. À titre d'exemple, dans le département de l'Essonne, des projets de téléphériques urbains entre les lignes C et D du RER ou à Paris-Saclay apporteraient des réponses efficaces aux déplacements en grande couronne dans l'attente de la très lente rénovation des RER, qui ne sera évidemment achevée que dans quinze

êtes-vous favorable à une remise à plat des grands projets d'investissements de transports dans notre région, seul moyen de réaliser plus de projets, plus rapidement, dans tous les territoires franciliens et avec des coûts moins importants

digitale, des nouvelles mobilités qu'elle rend possibles, de la fluidité qu'elle permet, dans des trajets qui associeront plusieurs réponses adaptées aux territoires,

Mme la ministre. Monsieur le sénateur, je ne peux pas laisser dire que la RATP s'est désintéressée de son réseau pour s'occuper du métro de Rio. Je tiens à rendre hommage à cette entreprise que je connais bien : elle a, avec détermination et constance, entretenu son réseau.

la RATP et la SGP -que le rythme des investissements doit être soutenable pour les transports de la vie quotidienne.

spécifique et remarquable. Je ne suis pas sûre qu'un big-bang de l'organisation en Île-de-France serait propice à une amélioration rapide des transports en Île-de-France.

des décennies de sous-investissement. Je comprends la règle de la priorisation sur l'entretien et la modernisation des réseaux pour les transports du quotidien, mais peut-être que toute bonne règle a son exception

plus forte croissance démographique, ainsi qu'une croissance économique exceptionnelle. La Seine-et-Marne produit un nombre de logements considérable. Elle participe de manière singulière à la création de valeurs et d'emplois dans la région. Or elle a toujours été la parente pauvre,

routières, interconnexions, développements et initiatives de transports nouveaux, notamment sur le réseau routier avec du matériel roulant sur les autoroutes.

Delouvrier et de Gaulle ont engagé voilà quarante ans le développement de l'Est francilien et de la région en général. Au-delà du plan d'investissement et de rénovation, nous avons besoin d'un nouveau Delouvrier pour préparer les investissements en infrastructures et en transports en commun.

doit avoir sa part des améliorations des transports. C'est le cas, par les schémas directeurs des RER, dans les programmes de régénération

-bénéficie non pas simplement aux habitants des territoires qu'ils desservent, mais bien à l'ensemble de la région. Cela suppose aussi de développer

L'État mettra à la disposition des autorités organisatrices et utilisera sur ses propres infrastructures toutes les innovations possibles, notamment pour développer le contrôle sanction automatisé, dédier des voies pour fluidifier la gestion du trafic

la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je suis usager de la ligne B, comme beaucoup d'entre vous ici, et je me rends régulièrement à Nanterre venant de de Bourg-la-Reine. À ce titre, j'ai l'immense plaisir d'emprunter les deux lignes les plus saturées d'Europe. C'est une souffrance, c'est quelque chose qui rend malade, au sens propre. Par ailleurs, n'est-il pas absurde

et aux problèmes d'organisation de la localisation du travail et de nos activités, il n'y a pas nécessairement des solutions techniques. Vous devez avoir une approche sociale des problèmes de transport.

à planifier le développement de la région sur les prochaines années en articulation avec le développement des infrastructures ; il s'agit d'un outil à la disposition des collectivités locales.

en claquant des doigts, alors que le sous-sol est l'un des plus compliqués qui existent au monde, et qu'on ne fait pas 36 milliards d'euros de lignes à grande vitesse sans en avoir les ressources. Nous traitons ces sujets avec beaucoup de détermination, d'engagement, de volonté d'améliorer les transports de nos concitoyens, mais aussi en faisant preuve de réalisme et de sincérité.

en région Île-de-France. Les Franciliens, peut-être plus que tous les autres habitants en France, ont souffert de la politique menée pendant des années et visant à donner la priorité au financement des lignes à

49 % sur les lignes de province et seulement 13 % dans le réseau francilien. Si l'on met en regard ces chiffres avec ceux de la fréquentation, on mesure davantage l'ampleur des difficultés.

élaborera avec détermination les programmes les plus efficaces pour permettre les résultats les plus rapides. Comme cela été remarqué tout à l'heure, on ne règle peut-être pas les problèmes en demandant des diagnostics sur les gares en Île-de-France, mais,

Réseau travaille avec beaucoup de détermination pour élaborer une stratégie d'investissement permettant des résultats visibles pour les voyageurs dans les meilleurs délais.

apportées par les contribuables franciliens depuis 2010- il faut rappeler que cela ne pèse pas sur le budget national

En effet, il est à craindre que la question du coût du Grand Paris Express, avec l'échéance des jeux Olympiques, donne lieu à un réarbitrage de certaines lignes, voire à une réalisation

la ministre, je souhaite avoir de votre part l'assurance que le projet du Grand Paris Express sera réalisé. Il en est de même pour la ligne 16, dont le Président de la République a parlé lorsqu'il est venu à Clichy-sous-Bois. D'un point de vue local, si je me réjouis de l'ouverture

Le Gouvernement est bien conscient des attentes fortes en matière de transport en Île-de-France, mais nous voulons sortir des calendriers irréalistes et des promesses non financées, pour proposer des trajectoires soutenables et crédibles. C'est dans cet

vont continuer à subir les retards et suppressions de train, à perdre leur emploi et à voir leur vie familiale se dégrader. Malheureusement, s'ajoute désormais au déséquilibre en matière d'investissements dans notre région une politique égoïste qui vise à exclure les voitures de Paris, sans augmenter simultanément et très sensiblement la qualité ou la quantité de l'offre de transports en commun pour les habitants de grande banlieue contraints de rejoindre la capitale pour des raisons

Est-il nécessaire de préciser que personne ne souhaite voir augmenter la pollution dans notre région ? Aussi, pourquoi certains feraient-ils semblant de croire que la pollution s'arrêterait aux limites du périphérique ?

c'est d'investir massivement pour l'amélioration des transports en grande couronne. Il est inacceptable que les recettes issues de la taxe du Grand Paris, payée par tous les contribuables de la région, bénéficient quasi exclusivement à la zone dense. On peut aussi s'interroger sur les recettes issues des vignettes récemment mises en place pour accéder à la capitale. Madame la ministre, êtes-vous favorable à un rééquilibrage significatif des investissements au niveau régional pour permettre la création, l'entretien, la modernisation et la transformation des réseaux de transports en grande couronne ? Très bien ! La parole est à Mme la ministre. Mme la ministre. Monsieur le sénateur, je pense que l'on ne peut pas opposer la grande couronne et la zone agglomérée ; on doit viser à réaliser les investissements qui permettront

bénéficient à l'ensemble des territoires, et pas uniquement à ceux qui sont traversés par l'infrastructure. Je suis convaincue que tel est bien l'objectif d'Île-de-France Mobilités : organiser la mobilité autour de ces infrastructures pour qu'elles bénéficient à l'ensemble des territoires d'Île-de-France. Pas du tout ! Je sais qu'Île-de-France Mobilités et les présidents des conseils départementaux ont beaucoup d'idées

qui étaient l'apanage de la région d'Île-de-France, sont en train de se développer dans toutes nos grandes métropoles. Il faut donc s'efforcer d'apporter des réponses rapides,

J'espère donc que, dans l'ordre des priorités que vous allez devoir établir, vous penserez à ces deux événements majeurs et que vous en tiendrez compte pour votre programmation. Nous avons attendu quarante-cinq ans la radiale entre Châtillon et Vélizy : nous aimerions bien ne pas attendre aussi longtemps

pas à la hauteur de ce qu'on pourrait souhaiter en Île-de-France, mais, en province, il n'y a pas de RER du tout : le réseau ferré national n'a pas été adapté pour tenir compte de l'émergence de nos métropoles. J'ai bien entendu

à la désaturation des réseaux ferroviaires dans les agglomérations, en Île-de-France, mais aussi en province, où le retard est également considérable.

S'il s'agit de créer un RER dans une grande ville de province qui n'en a pas, vous imaginez le délai ... Il va bien falloir qu'on trouve des solutions pour améliorer rapidement la mobilité de nos concitoyens, partout en France ! La parole est à M. Arnaud de Belenet,

c'est bien là la volonté de l'État. Les habitants de Seine-et-Marne paient la taxe sur le Grand Paris, comme tous les contributeurs franciliens, mais

la mobilité de nos concitoyens, vous avez raison de souligner que l'accueil des touristes, avec les grandes destinations qui se trouvent en Île-de-France, est aussi un enjeu important. Les opérateurs y travaillent, notamment fournissant des applications multilingues. Les offices de tourisme s'efforcent aussi de proposer des titres de transport.

d'une présence de la Brigade des réseaux franciliens, du renforcement des services de sécurité internes des opérateurs SCNF et RATP, de la présence humaine de ces opérateurs et de tous les outils modernes qu'on peut développer, notamment en matière de vidéoprotection.

tirer le meilleur parti d'un réseau de vidéosurveillance étendu. Il faudra continuer à travailler dans ce domaine, et le Gouvernement accompagnera les autorités organisatrices, en particulier Île-de-France Mobilités, pour aller dans ce sens.

en 2016 par l'État et la présidente de la région, Valérie Pécresse. Le pass Navigo à tarif unique a été instauré en 2015, sur l'initiative de Jean-Paul Huchon, à un prix de 70 euros, identique pour l'ensemble des Franciliens. En 2016, Valérie Pécresse, bien qu'elle ait promis pendant la campagne de ne pas augmenter le prix du pass Navigo, a engagé un bras de fer avec le Gouvernement, menaçant d'augmenter le prix à 80 euros ou 85 euros, sauf si l'État s'engageait sur un financement de l'ordre de 300 millions d'euros. Elle a alors conclu avec le Premier ministre un accord sur le financement du STIF, prévoyant notamment une augmentation de la taxe régionale sur les carburants, une hausse de la contribution pour les entreprises de la petite couronne de plus de onze salariés et une hausse du versement transport. Un an plus tard, le compte administratif de la région a pourtant révélé 300 millions d'euros non consommés dans le budget régional. Parallèlement,

Avec le recul, madame la ministre, diriez-vous que les sommes que la présidente de région a exigées de l'État n'étaient finalement pas justifiées,

les voyageurs en payant moins de 30 %. En Île-de-France comme ailleurs, on assiste à une baisse de la part payée par les voyageurs sur longue période ;, elle a diminué de dix points en dix ans. Cela pose la question de la soutenabilité du modèle, dans un contexte où personne personne n'imagine que les ressources des collectivités territoriales sont infinies- ou, pour le dire autrement, où chacun connaît les tensions qui existent sur les ressources publiques.

Je ne suis pas sûre que cela soit incompatible avec des tarifications solidaires, comme il s'en développe dans un certain nombre de métropoles en province,

il faudra aussi réfléchir à la façon dont chacun peut contribuer au développement des transports publics. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour le groupe Les Républicains.

Ce n'est pas une petite somme, j'en conviens, mais ce n'est pas un problème technique ; c'est une affaire financière. Il faudra donc que nous ayons des éclaircissements sur ce qu'on fait les uns et les autres pour arriver à de telles conclusions.

le RER A est toujours un élément disqualifiant de la vie quotidienne des habitants. Malgré les investissements de la région dans de nouvelles rames, malgré un schéma directeur de travaux de requalification, la nouvelle grille horaire mise en oeuvre en décembre dernier acte une baisse du nombre de trains, tout au moins au regard de l'offre théorique précédente. Aujourd'hui, à l'heure de pointe du matin, il est fréquent à Cergy-Préfecture de monter dans un train dont toutes les places assises sont occupées, alors qu'il y a encore sept arrêts avant La Défense.

un train bondé, en gare de Nanterre-Préfecture, gare de relève entre les conducteurs SNCF et RATP, sans un mot d'explication dans les haut-parleurs du train- je ne parle même pas d'excuses Si les inévitables aléas liés aux colis suspects ne peuvent être évités, ni négligés, les retards dus à des pannes techniques du réseau restent encore fréquents, quand on n'assiste pas à un arrêt total de la desserte pour cause de travaux mal dirigés pour EOLE. depuis toujours, la branche de Cergy, avec près de 50 000 voyageurs par jour, subit une iniquité insupportable quand elle se compare à la branche de Poissy- autant de RER par jour pour les 9 000 voyageurs de Poissy que pour les 50 000 de Cergy -et à celle de Saint-Germain-en-Laye- deux fois plus de RER pour pour à peine plus de voyageurs que sur la branche de Cergy. Madame la ministre, ma question porte donc sur l'état d'avancement des travaux sur le RER A : quand la SNCF et la RATP auront-elles enfin rattrapé trois décennies de sous-investissement ?

si les améliorations de l'infrastructure et le rattrapage de décennies de sous-investissement prennent du temps, les voyageurs peuvent heureusement voir les matériels financés par Île-de-France Mobilités, qui changent tout de même la vie, même si l'objectif est évidemment qu'ils roulent sur des infrastructures robustes robustes et fiables. Je ne suis pas en mesure de me prononcer, vous l'imaginez, sur la répartition des dessertes entre Poissy et Cergy et entre cette branche et celle de Saint-Germain-en-Laye.

Bon nombre d'orateurs ont souligné que le choix du tout-TGV, en absorbant les capacités d'investissement, a fait prendre un retard considérable dans la modernisation du réseau des transports franciliens, qui véhicule pourtant plus de passagers quotidiens que l'ensemble de nos lignes nationales. Avec le Grand Paris Express, une dynamique a été enclenchée en Île-de-France pour relier un certain nombre de territoires périphériques sans passer par Paris. Résultat d'un accord historique entre l'État et les collectivités territoriales, le Grand Paris Express, entièrement financé par des ressources exclusivement apportées par les contribuables franciliens, porte une ambition de développement sans équivalent. Cet engagement doit être tenu ! Ses atouts ? Desservir les territoires de petite et, en partie, de grande couronne- je pense aux lignes 16, 17, 18 et au Barreau de Gonesse, portes d'entrée dans la métropole qui complètent une offre de transports défaillante dans des territoires souvent socialement défavorisés. Ouvrir à l'urbanisation partielle et à l'aménagement des réserves foncières : triangle de Gonesse, plateau de Saclay, environnement de Roissy - Charles-de-Gaulle. Favoriser le développement économique en reliant les et en confortant de véritables pôles de compétitivité, tout en améliorant l'accessibilité des emplois. Si nous voulons que ce nouveau réseau soit pleinement efficace et tout simplement utile, la mise en connexion avec les lignes déjà existantes est fondamentale. Nous ne pouvons pas, madame la ministre, dépenser des milliards pour réaliser un manège forain en double boucle, que les usagers des transports urbains d'Île-de-France, singulièrement

Je pense particulièrement aux gares d'interconnexion, par exemple, pour la Seine-et-Marne, celles de Vert-de-Maisons et Bry-Villiers-Champigny avec la future ligne 15.

Leur défaut de financement, et donc de réalisation, serait très préjudiciable aux habitants de la grande couronne, qui seraient exclus de fait de ces nouvelles modalités de transports, alors qu'ils en sont financeurs, jusqu'à La Ferté-Alais, Château-Landon, Houdan ou Magny-en-Vexin. Cela n'est pas acceptable ! Madame la ministre, le précédent gouvernement avait pris de sérieux engagements pour que les deux gares d'interconnexion que j'ai citées soient réalisées en même temps que les travaux du Grand Paris Express. Pouvez-vous nous indiquer vos intentions sur ce point ? La parole est à Mme la ministre.

Comme vous le savez, il y a des débats entre l'État et la région sur le mode de financement de cette dernière interconnexion. En tout cas, pour ne pas retarder pour ne pas retarder et mettre en péril la réalisation de ces gares d'interconnexion, les études ont été engagées, ce qui permettra à l'État de poursuivre la discussion

Mme la ministre. Monsieur le sénateur, tout d'abord, je voudrais rappeler que les transports en Île-de-France sont totalement décentralisés. La responsabilité des transports est en effet confiée depuis maintenant de nombreuses années au Syndicat

Cette ligne est donc vitale pour près de 420 000 habitants ! Le Président de la République a rappelé à plusieurs reprises la nécessité que ce dernier tronçon soit dans la continuité de la tranche Le Bourget RER - Charles-de-Gaulle terminal 2, ou que l'ensemble des infrastructures soient finalisées dès 2025. La ligne 17 sera la garantie d'une certaine cohérence dans le réseau du Grand Paris Express. je vous rappelle avec insistance que la réalisation de ce réseau est envisagée pour l'accueil des jeux Olympiques en 2024. Or la Cour des comptes fait part aujourd'hui de sérieuses interrogations sur la capacité à respecter les échéances olympiques. Il me semble donc inenvisageable de sacrifier cette ligne au profit du projet CDG Express dont le but unique est de relier l'aéroport de Roissy à Paris. Ce projet reviendrait à abandonner la France des mobilités quotidiennes au profit des mobilités internationales.

Le métro du Grand Paris Express sans ces interconnexions amplifierait les écarts de croissance, de développement économique et urbain entre petite et grande couronne. Et cela, nous ne pouvons l'accepter

d'euros investis dans le réseau ferré national en Île-de-France, nous allons tripler le montant consacré à la modernisation du réseau par rapport à ce qui se faisait il y a une dizaine d'années. rappeler que le schéma d'ensemble du Grand Paris n'est pas remis en cause et que l'on doit travailler sur un phasage réaliste. Je souhaite enfin redire la volonté du Gouvernement de s'engager sur des calendriers crédibles,

CDG Express n'est absolument pas en concurrence avec les projets Ce projet qui ne bénéficie d'aucune subvention mais d'un prêt du Trésor public n'est en concurrence avec aucun des investissements dont nous avons parlé jusqu'à présent. Et l'entretien

Au Moyen Âge, la voie romaine Beauvais-Chartres desservait déjà la ville de Gisors dans l'Eure. Aujourd'hui, la voie romaine a disparu, les Capétiens et les Plantagenêts ne se mènent plus une guerre acharnée et Gisors est devenue une ville de près de 12 000 habitants. La question des transports reste un élément essentiel et central pour son développement. Gérée par Île-de-France Mobilités, la ligne J du réseau francilien dessert plusieurs villes de l'Eure, notamment Gisors et Vernon. La ligne J est en crise. Pour préparer mon intervention, j'ai échangé avec Alexandre Rassaërt, maire de Gisors, afin de faire un point précis sur la situation de cette ligne.

Les nouveaux horaires mis en place depuis le mois de décembre dernier, censés améliorer la ponctualité et la fréquence des trains, n'arrangent rien à la situation et ne font que l'empirer. La ligne J voit passer chaque jour près de 110 000 voyageurs, dont 1 300 Gisorsiens qui, pour beaucoup, ont fait le choix de s'installer en Normandie pour une raison simple : la proximité de Paris, leur lieu de travail. Imaginez la difficulté que cela engendre pour ces usagers à qui l'on avait promis un réseau de transport de qualité, gage de développement, qui permettrait d'attirer particuliers et entreprises dans cette belle région qu'est le Vexin normand. Pire, il semble que les élus des villes et communes hors de l'Île-de-France soient purement et simplement méprisés par les services chargés de gérer le réseau de transports. Le manque de considération à leur égard ne fait que renforcer un sentiment d'abandon de la province bien présent chez nos élus : celui du sacrifice des gares normandes sur l'autel des intérêts franciliens Madame la ministre, ma question est simple : comment comptez-vous améliorer la desserte des villes hors de l'Île-de-France par le réseau de transports francilien

en lien avec les régions qui peuvent aussi être en charge des TER dans leur périmètre. Ce que je peux vous assurer, madame la sénatrice, notamment les expertises de la Commission nationale du débat public ou les méthodes de concertation au service des autorités organisatrices pour s'assurer que les choix qui sont faits

Désignation des trente-sept membres du groupe de travail préfigurant la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance. Débat sur les conclusions du rapport d'information À seize heures trente : débat